La séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Les inégalités sociales jouent bien sûr un rôle important dans ces disparités. Mais les inégalités inhérentes au travail et à certains métiers sont tout aussi critiques. Les femmes ont tendance à travailler dans des secteurs à faible rémunération. Elles sont sous-représentées dans les postes de direction. Elles sont par ailleurs soumises à une pression plus importante visant à interrompre leur carrière pour des raisons familiales. Tous ces facteurs contribuent donc à creuser l'écart de revenus entre les sexes. C'est pourquoi il est essentiel que nous intégrions une approche par métier dans l'analyse comparative de genre menée par le Comité de suivi des retraites (CSR). Nous avons besoin d'une analyse approfondie des écarts de rémunération entre les sexes dans les différents secteurs et professions. Cela nous permettra de mieux comprendre les causes sous-jacentes de ces écarts et de formuler des recommandations pour les réduire. Madame Poncet Monge, celui entre les retraites des femmes et les retraites des hommes est encore plus élevé, comme nous le savons. En moyenne, la pension des hommes est de 39 % plus élevée que celle des femmes. Ainsi, la pension de droit direct

Cet écart est ainsi encore plus grand que l'écart entre les salaires, notamment parce que le montant de la retraite- un droit individuel -reflète que les femmes ont plus souvent que les hommes des interruptions de carrière, pendant lesquelles, si elles n'ont certes que pas

l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle a été étendue aux artisans et commerçants en 1972. L'objet de cet amendement est d'étendre cette majoration aux professionnels libéraux et aux avocats. Si les professionnels libéraux bénéficient de régimes autonomes adaptés à leurs spécificités ils ont bénéficié, au fil du temps, de l'harmonisation progressive des règles de leur régime de base avec celles du régime général. Cette harmonisation concerne notamment les règles de durée d'assurance, les pensions de réversion ou bien les majorations de durée pour enfant. Pour autant, les professionnels libéraux et les avocats ne bénéficient pas de la majoration de 10 % du montant de la pension pour trois enfants ou plus. mes chers collègues, c'est un dispositif de solidarité essentielle dans le panorama des droits familiaux de retraite. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales demande depuis plusieurs années que les professionnels libéraux

Pour autant, si les salariés, les artisans et les commerçants bénéficient de cette majoration, les professions libérales sont exclues de ce dispositif. Le 1février dernier, devant la délégation aux droits des femmes de l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, vous vous étiez dit ouvert pour avancer avec les parlementaires sur le sujet. Dans la foulée, le Gouvernement et plusieurs députés déposaient des amendements visant à étendre la majoration de 10 % de la pension pour trois enfants ou plus aux professions libérales. Malheureusement, les débats n'ont pas permis l'examen de ces amendements en séance publique. Dans une démarche de remise à niveau de la protection sociale des professions libérales, notre amendement prévoit d'étendre cette majoration aux professionnels libéraux et aux avocats. C'est une question d'équité. Il est en effet injuste que ces professions soient exclues de ce dispositif alors qu'elles contribuent au financement de cet avantage par le biais des cotisations d'allocations familiales, de la contribution sociale

profession d'avocat et à l'ensemble des professions libérales. Au préalable, je note que, contrairement au projet de 2019, votre gouvernement, monsieur le ministre, s'était engagé à ne pas toucher au régime autonome de retraite des professions libérales, dont celui des avocats. La profession, dont la mobilisation à la fin de 2019 et au début de 2020 avait été historique, le vit comme un soulagement, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Nous appelons à entendre la mobilisation qui s'exprime actuellement chez celles et ceux qui sont concernés. Le monde de la justice, vous le savez, souffre actuellement d'un sous-investissement, de délais de traitement interminables qui mettent à mal les justiciables et démotivent l'exercice de la défense. C'est dans ce contexte que je vous propose d'adopter cet amendement permettant d'aligner le régime des majorations de pension pour les parents de trois enfants et plus. Cette majoration est assurée financièrement par la caisse d'allocations familiales (CAF), abondée par les cotisations sociales des avocates et des avocats, qui, pourtant, ne peuvent prétendre à cette majoration de pension. Au lendemain de nos débats sur la compensation des temps familiaux, et après avoir entendu le discours défendant la valeur famille sur ces travées, j'imagine que vous ne pourrez que voter cet amendement, dont le financement est assuré par les bénéficiaires, à hauteur de 100 millions d'euros, par le biais des cotisations familiales,

présenter l'amendement n° 48 rectifié. Cet amendement a le même objectif que l'amendement que j'ai défendu précédemment. Il s'agit de permettre aux professionnels libéraux de bénéficier de la majoration de 10 % du montant de la pension pour trois enfants ou plus, à l'instar de ce qui existe déjà pour les salariés, les artisans et les commerçants.

par l'ordonnance du 19 octobre 1945. Elle a été étendue aux artisans et commerçants en 1972. Il s'agit ici d'étendre cette majoration aux professionnels libéraux.

ils ne bénéficient toujours pas de la majoration de 10 % du montant de la pension pour trois enfants ou plus. Or c'est un dispositif de redistribution horizontale essentiel. La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) le demande depuis plusieurs années, avec raison.

commencés après le 1 janvier 2012 fussent désormais prises en compte dans le salaire de base. Jusqu'en 2010, ces indemnités journalières étaient seulement prises en compte au titre de la durée d'assurance requise. Or le salaire de base et la durée d'assurance ont leur importance dans le calcul de la pension. Cette réforme n'était pas allée au bout de la logique, ne s'appliquant pas aux femmes ayant eu des enfants avant le 1 janvier 2012. L'amendement que je vous présente permet d'ouvrir cette possibilité à celles qui partiront à la retraite à compter du 1 septembre 2023. Si le montant des indemnités journalières versées n'est plus connu, le calcul pourra tenir compte d'un montant forfaitaire en rapport avec le montant des indemnités journalières dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé maternité.

C'est pourquoi cet amendement prévoit, pour les retraites liquidées à partir du 1 septembre 2023, de prendre en compte les congés maternité. Il permet d'ouvrir cette possibilité pour celles qui partent à la retraite à compter du 1 septembre 2023. Si le montant de l'indemnité journalière versée n'est plus connu, le calcul pourra donc tenir compte d'un montant forfaitaire, par exemple en rapport avec le montant des indemnités journalières dont peut bénéficier un salarié rémunéré au niveau du salaire médian l'année précédant le congé maternité. C'est une mesure de justice à l'égard des femmes, particulièrement celles qui sont en bas de l'échelle des salaires, lesquelles verront le montant de leur pension augmenter en fonction du nombre d'enfants qu'elles ont eus, les trimestres de maternité étant ainsi neutralisés. Cette mesure

l'amendement n° 3414. Prenant en compte l'inégalité que peuvent subir les femmes qui ont eu des enfants, la loi du 9 novembre 2010 avait prévu que les indemnités journalières versées dans le cadre des congés maternité commencés après le 1 janvier 2012 soient désormais prises en compte dans le salaire de base, et non uniquement- il faut le souligner -au titre de la durée d'assurance requise servant au calcul de la pension. Cependant, cette réforme n'était pas allée au bout de sa logique, puisqu'elle ne s'appliquait pas aux femmes ayant eu des enfants antérieurement au 1 janvier 2012. Cela est malheureusement assez peu compréhensible et constitue, une nouvelle fois, une injustice envers les femmes qui n'a que peu de fondement. Dès lors, cet amendement vise à revenir sur ces dispositions et à permettre que les indemnités journalières des femmes avec enfants soient prises en compte dans le salaire de base servant au calcul de la pension. Dans le cas où le montant d'indemnités journalières versées n'est plus connu, il est alors tenu compte d'un montant de base qui est celui dont peut bénéficier une salariée rémunérée au niveau du salaire médian l'année précédant le congé maternité. Cela semble une idée raisonnable, voire de bon sens. En conséquence, je salue l'avis favorable de la commission et espère l'adoption d'un amendement qui ne peut qu'améliorer la situation de nombreuses femmes dans le pays. Quel est l'avis de la commission ?

collègues, la situation dans ces territoires est particulièrement dégradée. Selon l'Insee, en 2020, 16 % à 23 % de personnes vivent sous le seuil de pauvreté local dans les outre-mer. Aux Antilles et en Guyane, une personne sur cinq vit en deçà du seuil de pauvreté local, qui est de 820 euros mensuels en Martinique et de seulement 550 euros en Guyane. En conséquence, la proportion de personnes ayant une pension faible et qui dépendent de l'Aspa est importante. Malgré tout, les sommes versées au titre de cette allocation sont récupérées au décès de l'allocataire au-delà d'un certain seuil. est non pas simplement injuste, mais également dissuasive ; et le non-recours est évidemment important. Dans le cadre d'une expérimentation menée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) visant à contacter les personnes éligibles à l'Aspa, les motifs de non-recours invoqués étaient la méconnaissance de la prestation et l'existence de cette fameuse récupération sur succession, de sorte que le taux de non-recours est de 50 %. Je crois que nous privons ici une partie importante de la population d'une aide non négligeable qui leur permettrait de vivre un peu plus dignement lors de leur retraite. De manière générale, la reprise sur succession n'a que peu de justification,

Il existe un certain nombre d'outils pour lutter contre cette pauvreté des retraités, comme l'Aspa. L'Aspa est une allocation versée aux personnes de 65 ans et plus ou aux personnes inaptes, sous condition d'un plafond de ressources qui dépend de la situation de la personne. Elle est versée par la caisse de retraite à laquelle la personne est affiliée. Il pourrait s'agir d'une allocation permettant effectivement de lutter contre la pauvreté des personnes de 65 ans et plus, mais elle est- on le sait -très mal connue en France.

seulement 325 700 d'entre elles sont effectivement bénéficiaires de l'Aspa. Le taux de non-recours de cette allocation se situe autour de 50 %. Une partie des potentiels bénéficiaires ne sont tout simplement pas au courant de l'existence de ce dispositif, même si celui-ci a été introduit il y a désormais dix-sept ans. D'autres hésitent à demander l'Aspa, car les sommes versées à ce titre sont récupérées au décès de l'allocataire sur sa succession si l'actif net successoral est au moins égal au seuil de recouvrement. Cette situation devrait nous interroger sur deux points : les potentiels bénéficiaires sont-ils suffisamment informés de leurs droits ? Les conditions d'accès sont-elles appropriées ? Il convenait de se demander notamment si la récupération des versements en cas de décès sous certaines conditions ne rebute pas des personnes potentiellement éligibles.

trop rares dans ce projet de loi : la possibilité de valider comme trimestres cotisés des périodes travaillées en stage de formation professionnelle, dont celles qui ont été effectuées dans le cadre des travaux d'utilité collective, pour les retraités partant après le 1 septembre 2023. J'évoque les travaux d'utilité collective parce que je pense que, sur l'ensemble des travées de cet hémicycle, nous avons reçu de très nombreux messages venant de salariés qui ont été des « tucistes » et qui nous ont sollicités sur la nécessité de remédier Mais, hélas ! je veux souligner que, comme souvent, vous n'allez pas au bout de vos avancées, alors que vous n'hésitez jamais à aller au bout de vos idées lorsqu'elles constituent une régression sociale, comme c'est le cas, bien entendu, du passage à 64 ans de l'âge légal de départ à la retraite. De qui parlons-nous ? Nous parlons de jeunes qui étaient âgés, dans les années 1980, de 16 à 25 ans, rémunérés à hauteur de 1 250 francs par mois et pris en charge par l'État. En fait, ces tucistes étaient des jeunes globalement plus précaires que la moyenne. Si vous n'assouplissez pas les règles applicables pour justifier l'existence d'un contrat, il est certain que de trop nombreuses personnes n'arriveront pas à faire valoir leurs droits. Je présenterai d'ailleurs un amendement en ce sens pour améliorer ce dispositif.

il n'avait pas été prévu que les trimestres de TUC effectués soient pris en compte pour la retraite. C'est pourquoi les anciens bénéficiaires de ce dispositif, qui partent désormais à la retraite, se sont mobilisés récemment pour obtenir gain de cause. Je veux saluer cette mobilisation ; comme cela a été dit, beaucoup d'entre nous ont été sollicités par par ces personnes, et nous avons aussi interpellé le ministre à ce sujet. Toutefois, il est regrettable de ne pas rendre rétroactive la validation de trimestres pour les personnes qui ont pris leur retraite avant le 1 septembre 2023. Alors que le Gouvernement chiffre le coût de cet article à moins de 100 millions d'euros une fois la montée en charge réalisée, et que seuls 5 % des assurés ayant effectué des TUC sont partis à la retraite, une telle rétroactivité ne coûterait pourtant qu'environ 5 millions d'euros par an.

mesure aux personnes qui prendraient leur retraite avant le 1 septembre 2023. Cet effet de seuil est particulièrement malvenu, vous en conviendrez.

à celui de la création de droits à retraite. En effet, les élus qui perçoivent des indemnités de fonction mensuelles inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale, soit 1 qui, par ailleurs, n'ont pas cessé toute activité professionnelle ne cotisent pas au régime de base de la sécurité sociale. Ils ne valident donc pas nécessairement quatre trimestres par an et leurs indemnités n'ouvrent aucun droit à retraite au régime de base. Plus de 80 % des maires, quasi exclusivement de communes de moins 4 000 habitants, sont potentiellement concernés. De surcroît, ils sont de plus en plus nombreux à réduire leur activité professionnelle pour exercer leur mandat. Pour leur permettre d'ouvrir des droits à retraite, cet amendement vise donc à offrir la possibilité aux élus locaux d'être assujettis aux cotisations de sécurité sociale, dont la cotisation d'assurance vieillesse, sur l'indemnité de fonction qu'ils perçoivent. Cette disposition s'exerce sur option par l'élu, donc de manière non obligatoire. Par ailleurs, tout assuré peut effectuer un versement pour la retraite au titre des années d'études supérieures et des années de cotisation incomplètes. Ces rachats de cotisations manquantes permettent de conforter et de sécuriser la pension de retraite des assurés. Ils sont limités à douze trimestres. Or l'actuel dispositif de rachat de trimestres étant ouvert pour les années incomplètes, il empêche le rachat de trimestres pour les années au cours desquelles un élu n'en aurait validé aucun. cet amendement tend également à ajouter les années de mandat électoral à la liste des situations permettant le rachat de trimestres. Je remercie M. le ministre, ainsi que Mme et M. les rapporteurs

que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous vous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien jusqu'au terme de

Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. C'est vous qui faites

d'amendement ! Comme les précédents, notre amendement vise à ouvrir la possibilité aux élus dont le montant total brut des indemnités de fonction est inférieur à 1 833 euros par mois

un droit à une retraite décente afin que ceux qui ont consacré de nombreuses années au service de leurs concitoyens ne soient pas pénalisés au moment de leur départ à la retraite.

et à combattre la crise des vocations constatée en ce domaine, particulièrement dans les petites communes. Retirez-le ... Nous savons tous que l'exercice d'un mandat local représente pour les élus une charge de plus en plus lourde sous l'effet conjugué de la poursuite des transferts de compétences de l'État vers les collectivités territoriales et d'exigences de plus en plus importantes. Quel

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas. L'amendement n° 2214

de la nécessité de conserver leurs documents administratifs, comme les bulletins de salaire ou les contrats de travail, pour justifier de leurs droits à la retraite. Or, dans la mesure où les TUC n'ouvraient aucun droit

: La parole est à M. Daniel Salmon. Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas.

L'État finançait la rémunération des TUC à hauteur de 1 200 francs, soit environ 180 euros- un quart du Smic d'alors -, pour 80 heures par mois. Or ils ne cotisaient pas assez pour permettre l'acquisition de trimestres pour leur retraite.

nous proposons qu'une simple attestation écrite de la structure au sein de laquelle les travaux ont été réalisés soit suffisante pour constituer un justificatif valable pour le calcul de la retraite. Quel

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées.

L'État se charge de payer les cotisations manquantes si la rémunération n'est pas suffisante. En revanche, du 1 juillet 1972 au 31 décembre 2013, la prise en compte n'est que partielle et le nombre de trimestres validés inférieur au nombre de trimestres d'apprentissage réalisé.

Votre objectif était sans doute que nous vous laisserions ensemble, les droites coalisées, décider de la retraite des Français. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus, et, à chacun de nos amendements, nous tenons à rappeler à ceux qui nous regardent que nous ne lâcherons rien et que nous ne les lâcherons pas.

validation rétroactive, pour le décompte de la retraite, les trimestres réalisés en tant qu'apprenti avant la réforme de 2014. Néanmoins, compte tenu de l'importance du sujet et de l'urgence pour les anciens apprentis concernés, il paraît souhaitable que le rapport soit remis avant onze

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien. » Les auteurs du

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. » C'est le même discours

nous n'avons plus beaucoup d'armes pour lutter contre cette réforme injuste parce que vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par la conjonction de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. C'est du comique de

rapport vise à estimer le coût et la faisabilité de valider rétroactivement, pour le décompte des droits à la retraite, les trimestres réalisés comme apprenti avant la réforme de 2014. Néanmoins, compte tenu l'importance du sujet et de l'urgence pour les anciens apprentis concernés, il paraît souhaitable que le rapport soit remis dans les dix mois qui suivent la promulgation

: vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien ; nous ne les lâcherons pas. Les Français regrettent la tournure que prennent nos séances, qui ne sont plus qu'un exercice de lecture de nos amendements, sans débat et sans vote.

pour le décompte de la retraite, les trimestres réalisés en tant qu'apprenti avant la réforme de 2014. Néanmoins, compte tenu de l'importance du sujet et de l'urgence pour les anciens apprentis concernés, il paraît souhaitable que le rapport soit remis avant onze mois après la promulgation de la loi.

Vous avez décidé d'abaisser »- je change un mot -« la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien.

change un mot -« la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien. » Les auteurs du

Pour celles et ceux qui ont été en apprentissage avant le 1 janvier 2014, cette réforme des retraites serait la double peine. En effet, jusqu'au 1 janvier 2014, les trimestres d'apprentissage n'étaient pas entièrement pris en compte pour les droits à la retraite. Heureusement, la réforme de 2014 est venue corriger ce problème, en permettant une validation automatique de tous les trimestres d'apprentissage. Cependant, la mesure n'a pas été rétroactive et n'a donc pas permis aux personnes ayant été en apprentissage avant 2014 de valider ces trimestres. Prenons l'exemple d'une personne née en 1968 et ayant commencé un apprentissage en 1987, quand elle avait 19 ans. Cette personne serait concernée par la présente réforme, alors qu'elle ne l'était pas par la réforme permettant la validation des trimestres en 2014. Elle est victime du relèvement de l'âge légal de départ, sans pouvoir faire valoir ses trimestres d'apprentissage. Puisqu'elle devra travailler plus longtemps après l'adoption de la réforme, il faudrait reconnaître ses trimestres d'apprentissage,

tôt pouvaient cotiser plus longtemps. Toutefois, cette réforme des retraites change complètement la donne, parce qu'elle repousse l'âge légal de départ et augmente le nombre de trimestres nécessaires. La justification que je viens d'évoquer ne tient donc plus. Cet amendement demande un rapport sur la faisabilité d'une validation rétroactive des trimestres des apprentis réalisés avant l'entrée en vigueur de la réforme de 2014. Je profite de mon intervention pour envoyer une petite salutation à Justin, un apprenti que je connais bien. Quel

monsieur le ministre,

d'intégrer les trimestres rachetés dans les trimestres pris en compte pour le départ anticipé au titre des carrières longues, puisque le rachat de trimestres prévu par la loi de 2014 n'autorisait pas leur intégration aux conditions d'éligibilité au dispositif de carrières longues et, donc, au départ anticipé. Nous avons pris l'engagement de faciliter l'information et les conditions de rachat de ces trimestres d'apprentissage, avec

de tous les procédés que vous fournissent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous escomptiez sans doute que nous abandonnerions la retraite des Français au soin des droites liguées. Nous ne sommes pas les dindons de la farce, les Français non plus. Nous ne flancherons pas ; nous ne les laisserons pas tomber.

je tiens à faire aujourd'hui une exception, car j'ai l'honneur, en solidarité avec tous mes amis des groupes de gauche, de vous dire que vous avez décidé de dévitaliser et d'anesthésier la fonction parlementaire, monsieur le président, par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien ; nous ne les lâcherons pas. Amen ! Cet amendement

votre état d'esprit, votre volonté d'agir, votre efficacité et votre tempérament, nous proposons que ce rapport soit remis au bout d'un an,

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous vous laisserions tranquillement entre vous décider de la retraite des Français.

le disait à l'école, mes chers collègues, vous recopierez cent fois ! Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous vous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous non plus ! Ils le montreront encore tout à l'heure. Pour notre part, nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas.

nous ne les lâcherons pas face à la crise politique et sociale qui se profile dans notre pays, nous ne les lâcherons pas face au risque populiste très grave qu'entraîne le passage en force de ce texte. Ce sous-amendement vise à renforcer l'amendement de notre collègue Éliane Assassi pour limiter le non-recours aux droits,

confine à l'obstruction, M. le rapporteur l'a dit. Il permet aussi de souligner que les dispositions prises par la conférence des présidents du Sénat, demandées par certains présidents de groupe et mises en oeuvre par le Gouvernement, relèvent de la Constitution et du règlement, ce qui témoigne de leur régularité.

Nous souhaitons que cette durée soit allongée. En effet, la durée moyenne d'inscription sur la liste de haut niveau, pour des sports comme l'athlétisme et l'aviron, se situant entre huit et dix ans, l'ouverture des droits sur quatre ans ne recouvre ainsi même pas la moitié d'une carrière internationale. Par

frères ... ... à mon tour, je vous le dis : vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus.

possible compensation par l'État des trimestres non cotisés par les sportifs de haut niveau en complétant, à hauteur de quatre trimestres par an, pour tous les régimes de retraite de base, les droits à pension de ces sportifs aux carrières extrêmement courtes. Afin que ce rapport ne reste pas lettre morte, ils souhaitent que soit expressément prévu, aux termes de la loi, que celui-ci fasse l'objet d'un débat dans les quatre commissions parlementaires des affaires sociales et des affaires culturelles.

il a jugé utile de nous rappeler que les procédures utilisées étaient légales. C'est bien le moins, monsieur le ministre ! J'espère que, si tel n'était pas le cas, l'indignation ne s'élèverait pas uniquement des travées de la gauche et serait partagée par la totalité du Sénat.

ou les sous-amendements n'ont pas été examinés par la commission. Moralité : si la commission des affaires sociales avait été réunie, il n'y aurait pas pu avoir ce vote bloqué. Je le dénonce, avec l'ensemble de mon groupe.

plus ! Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions les retraites des Français entre les

? -sur la possibilité de rendre rétroactive la validation comme trimestres cotisés de périodes travaillées en stage de formation

vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement Vous espériez que nous laisserions les retraites des Français aux mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus.

En conséquence, il apparaît que les trimestres chômés, à l'instar des trimestres travaillés, sont,, mieux pris en compte que le choix de faire une formation professionnelle,

dans le calcul des droits à la retraite. Entre 1985 et 1990, l'État a employé plus de 350 000 personnes sous contrat « TUC ». Âgés de 18 à 20 ans, les chômeurs de l'époque ont accepté des missions de service public afin de ne pas être radiés

professionnelle ; de ce fait, cette période n'est pas comptabilisée dans le calcul de leurs droits à la retraite. Grâce à leur mobilisation sans faille et au travail d'un certain nombre de parlementaires, ils ont obtenu gain de cause. C'est une avancée positive. Ils n'ont rien lâché, et nous non plus Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions les retraites des Français entre les mains des droites coalisées ; nous ne sommes pas dupes, les Français non plus ! Nous ne lâcherons rien,

Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement.

Afin que ce rapport ne reste pas lettre morte, nous souhaitons que soit expressément prévu, aux termes de la loi, qu'il fasse l'objet d'un débat dans les deux commissions parlementaires des affaires sociales. L'amendement

sorte la double peine. Cet amendement a donc pour objet de demander à la Cnav un rapport sur la possibilité de rendre rétroactive la validation comme trimestres cotisés des périodes travaillées en stage de formation professionnelle, dont celles qui le furent dans TUC. Le texte ne prévoit une telle validation que pour les personnes partant à la retraite à partir du 1 septembre 2023. Il me reste un peu de temps ; je voudrais donc marteler une fois de plus, pour que nul ne l'ignore, que vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de tous les procédés que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas ! l'avis de la commission

que nous laisserions la retraite des Français entre vos mains, celles des droites coalisées. Mais nous ne sommes pas dupes, et les Français non plus ; ils vous le rediront cet après-midi. Nous ne lâcherons rien, comme eux ne lâcheront rien ! Voilà ce qu'inlassablement nous voulons vous dire, amendement après amendement.

Ne nous leurrons pas : si le Gouvernement a décidé de reprendre les dispositions préconisées par la mission flash de nos collègues députés, cela n'atténue en rien l'injustice de cette réforme.

de pouvoir prendre leur retraite. Une proposition de loi sur les droits des bénéficiaires des TUC était pourtant prête et aurait pu être choisie comme véhicule législatif sans passer par cette injuste réforme des retraites. Tel est l'objet de notre amendement

(SMA), dispositif d'insertion socioprofessionnelle prévu au bénéfice exclusif des jeunes de 18 à 25 ans éloignés de la qualification et de l'emploi et résidant dans les outre-mer. Le SMA peut accueillir chaque année 6 000 bénéficiaires, dont 60 de non diplômés et environ 40 % de jeunes illettrés, selon la catégorisation de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Il permet de suppléer au déficit de structures dans le domaine de la formation professionnelle des jeunes dans les outre-mer et constitue aujourd'hui un dispositif important et reconnu par les employeurs locaux pour sa qualité et son efficacité

Vous avez en effet décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas

Mme Sabine Van Heghe. Les trois groupes de gauche déplorent l'attitude du Gouvernement qui, avec la complicité « naturelle » de la droite sénatoriale, fait passer en force sa réforme des retraites en utilisant la procédure de vote bloqué sur des amendements déjà choisis- aucun des nôtres, Oui, monsieur le ministre, mes chers collègues de la majorité sénatoriale de droite, vous avez décidé de vider de son sens la fonction parlementaire grâce à toutes les procédures offertes par la Constitution et par le règlement du Sénat.

demander la remise d'un rapport sur l'impact de la réforme de la liquidation unique des régimes alignés sur les travailleurs transfrontaliers. Nous sommes en effet saisis de nombreux cas d'assurés qui, travailleurs transfrontaliers, se voient lésés par la mise en oeuvre de la réforme. En effet, il semble que les caisses de retraite n'appliquent plus de proratisation sur la durée d'assurance dans la sélection des meilleures années pour le calcul du salaire annuel moyen de référence, comme ce fut le cas jusqu'en juillet 2022 pour les travailleurs frontaliers. Cela conduit à retenir dans la formule de calcul du salaire annuel moyen

s'agir également de l'année au cours de laquelle l'assuré est parti à l'étranger, et pour laquelle le revenu annuel français est donc particulièrement faible. Puisque ces années tirent ensuite le salaire annuel moyen vers le bas,

À cette fin, il suffirait par exemple de calculer le salaire annuel moyen sur la base de 60 % des « meilleures » années travaillées en France. En d'autres termes, au lieu d'utiliser un nombre absolu d'années, le nombre d'années prises en compte serait proratisé en fonction de la durée de la carrière française.

par année civile. Nous non plus, nous ne lâchons pas les Français

du public ; cet engagement les honore. Ils ne lâchent pas la population et nous ne les lâcherons pas non plus, même si vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas. Et nous ne lâcherons pas, en l'espèce, nos sapeurs-pompiers volontaires. Nous demandons donc une majoration de leur durée de cotisation une bonification de trois

Tout l'été, des milliers de pompiers volontaires et professionnels se sont battus contre les flammes à travers la France. Des renforts de pompiers grecs, autrichiens ou allemands ont même été nécessaires. Il faut donc que nos pompiers soient plus nombreux

regrettable que vous ayez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Pas vous ! Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées, mais nous ne sommes pas dupes,

de la Nation que tout le monde ici soutient avec force et vigueur.

mais une indemnisation exonérée de tout prélèvement social. Les sapeurs-pompiers bénévoles ne cotisent donc pas pour leur retraite, et aucun trimestre ne peut leur être alloué à ce titre. Pourtant, les sapeurs-pompiers volontaires, tout comme les professionnels, interviennent dans le cadre d'opérations de secours à des personnes, de protection des biens et de l'environnement, d'extinction des incendies. Cette activité bénévole présente de forts risques pour la sécurité et la santé des personnes qui s'y engagent. Surtout, les services départementaux d'incendie et de secours seraient réduits à peu de chose sans les sapeurs-pompiers volontaires. En effet,

plus là-dessus que sur le reste. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées ; vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de tous les procédés que vous offrent la Constitution et notre règlement. Les Français ne sont pas dupes, nous non plus : nous ne les lâcherons pas

entre vous, à droite, ensemble. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne lâchons rien et nous ne lâchons pas les Français, qui se mobiliseront massivement cet après-midi ! L'article 12, en essayant de faire passer la pilule de cette loi scélérate, s'intéresse aux aidants. C'est commode, les aidants. C'est comme la carte au jeu des Mille bornes : on la sort quand on est manifestement bloqué et que l'on veut avancer. Votre gouvernement a joué cette carte, monsieur le ministre, lors de la réforme du marché du travail.

cette réforme a profondément modifié la VAE dans tous les secteurs professionnels. Les aidants étaient déjà un prétexte. Doit-on voir dans cette autre chose qu'un prétexte pour repousser l'âge de la retraite ? Je le pense. Les critiques entendues le confirment : cela existait déjà, on ne part pas de rien, l'assurance vieillesse du parent au foyer existe, mais son accès est très restrictif.

porteur de handicap et qui perçoivent une allocation d'éducation pour enfants handicapés. Pourquoi ne pas maintenir les droits à la retraite sur cette base ?

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien et, surtout, nous ne lâcherons pas les Français

11 millions de nos concitoyens prennent en charge des enfants et des personnes handicapées, qu'ils soient très proches ou plus éloignés.

Enfin, je voudrais dire à notre collègue Patriat, qui a dû s'absenter, que, si nous sommes minoritaires au Sénat, en revanche, nous sommes majoritaires dans le pays.

qui tente de maquiller l'injustice de votre projet de loi et le piétinement de nos acquis sociaux. Certes, cet article, qui traite du régime de retraites des aidants familiaux, permet l'élargissement du périmètre de l'AVA à certaines situations non prises en compte. Mais

Car nous le savons toutes et tous, il est déjà possible pour la plupart des aidants de valider des trimestres de retraite, qu'il s'agisse de parents d'enfants en situation de handicap ou de proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie. La seule avancée permise par cet article est l'éligibilité à la validation de trimestres des parents qui sont bénéficiaires d'un complément

par exemple les deux membres d'un couple. C'était d'ailleurs l'objet de notre amendement n° 4589, déclaré irrecevable. Les associations demandaient aussi l'affiliation à l'AVA de tous les parents d'un enfant en situation de handicap ou la possibilité pour les aidants de partir à taux plein avant l'âge légal. Comme pour tant d'autres mesures utiles, attendues par nos concitoyens, porteuses de justice sociale, il n'en sera rien : elles sont balayées parce que vous avez décidé de de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains d'une droite coalisée. Il faut conclure ! Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus ! Nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas

l'article 12 est particulièrement important puisqu'il prévoit une nouvelle mesure pour la reconnaissance des aidants familiaux. Cet article a en effet pour objet la création d'une assurance vieillesse pour les aidants familiaux à laquelle seraient affiliés les actuels bénéficiaires de l'assurance vieillesse des parents au foyer, qui assument la charge d'un enfant ou d'un proche handicapé. Il vise à étendre l'affiliation de ce dispositif à de nouveaux bénéficiaires. Ainsi, les personnes bénéficiant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé auront droit à l'AVA. Cette disposition permettra de compenser la réduction d'activité d'un des parents du fait du handicap d'un enfant dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 70 %. Mes chers collègues des travées de gauche, vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par toutes les procédures à votre disposition pour « emboliser » les débats. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus ! Les gauches coalisées par leur obstruction ne veulent ni débattre ni voter ! Au contraire, nous souhaitons aller jusqu'au bout de ce projet de loi pour garantir une retraite à nos concitoyens.

Merci

Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien, et nous ne les lâcherons pas Depuis le début de l'annonce de cette réforme des retraites, le Gouvernement multiplie les mensonges. Nous avons précédemment pu évoquer les 1 200 euros pour tous les retraités, mais ce n'est qu'un des nombreux mensonges de ce gouvernement. Nous pouvons en citer un autre : le fait que cette réforme serait équitable, porteuse de justice et de progrès social. En réalité, personne n'est dupe : contrairement à ce que vous affirmez ce que vous affirmez partout, cette réforme fera évidemment des perdants. Cette réforme fait porter encore l'effort sur les femmes. Aujourd'hui, elles partent déjà plus tard à la retraite et touchent des pensions plus faibles que les hommes. Avec votre réforme, elles seront davantage touchées par le report de l'âge légal : sept mois de

quatre pour les hommes de la génération de 1980. C'est inadmissible ! Alors que la situation des femmes est déjà compliquée puisque 40 % d'entre elles partent à la retraite avec une carrière incomplète et que 20 % attendent attendent l'annulation automatique de la décote à 67 ans pour partir à la retraite, contre 10 % pour les hommes, votre réforme va aggraver cette situation au lieu de l'améliorer. Tous ces mensonges nous poussent à proposer cet amendement pour associer le Conseil d'État à l'écriture des décrets. Car ce gouvernement n'est pas digne de confiance et méprise le peuple français en bâillonnant le Parlement avec l'article

Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas ! Nous avons pu, depuis le début de l'examen cette réforme, citer les nombreux mensonges et incohérences de ce gouvernement, qu'il s'agisse de l'impact de la réforme sur la retraite des femmes, de la retraite à 1 200 euros pour tous ou de son caractère inéluctable. Autre argument argument entendu en boucle dans toutes les interviews depuis le 10 janvier : le problème démographique que connaîtrait notre pays rendrait cette réforme obligatoire pour sauver notre système de retraite par répartition. ratio entre les actifs et les retraités s'est effectivement réduit, puisqu'il est passé de 3 actifs par retraité à 1,7 actif par retraité, notre système a continué à tenir solidement, notamment grâce à une hausse des cotisations payées par ces mêmes

Cette réforme révèle donc deux choses importantes. Premièrement, elle révèle que le Gouvernement refuse de soutenir la hausse des salaires et leur indexation sur l'inflation alors que cela permettrait de résoudre en grande partie le problème du futur déficit du système de retraite. que vous avez abandonné l'idée d'une accélération de la productivité alors même que toutes les aides et exonérations de cotisation que vous offrez aux entreprises ont justement pour but d'accélérer cette productivité.

souhaitent que les décisions réglementaires en matière d'incapacité d'enfant ou d'adulte nécessitant la présence d'un aidant qui puisse avoir des droits soient accompagnées d'un éclairage des instances représentatives des personnes en situation de handicap. Selon le baromètre 2017 de la Fondation April et de BVA, 11 millions d'aidants familiaux, soit un français sur six, accompagnent au quotidien un proche en situation de dépendance en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. Ces chiffres sont en constante augmentation. L'affiliation à l'assurance vieillesse pour les aidants permet à l'aidant familial de valider des trimestres pour sa retraite sans qu'il ait besoin de verser des cotisations auprès de sa caisse de retraite. Des diagnostics largement convergents montrent qu'il est nécessaire de mettre en place un véritable statut du proche aidant, qui lui confère un certain nombre de droits, plus complets et mieux identifiés, parmi lesquels des droits revus en matière de cotisation à la retraite. Il s'agirait notamment de revoir quel taux d'incapacité permanente d'un enfant ou d'un adulte nécessite son accompagnement au quotidien par des aidants. C'est pourquoi, dans un souci de plus grande justice sociale concernant ces situations, les auteurs de cet amendement proposent que ces taux d'incapacité soient fixés certes par décret, mais après consultation des instances représentatives des personnes en situation de handicap. Je crains néanmoins que nous ne puissions pas voter cet amendement, car vous avez décidé dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas

pour présenter l'amendement n° 772 rectifié. En France, 8 à 11 millions de personnes soutiennent au quotidien un proche en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Ces aidants sont bien souvent conduits à interrompre leur carrière professionnelle, ce qui a un impact sur les droits à la retraite, du fait d'une interruption ou d'une réduction de leur activité. Aujourd'hui, l'assurance vieillesse des parents au foyer permet de prendre en compte, au titre de l'assurance vieillesse, les périodes d'interruption ou de réduction de l'activité professionnelle consacrée à l'éducation des enfants ou à la prise en charge d'un proche en situation de handicap ou en perte d'autonomie. Ce dispositif souffre toutefois d'un défaut de lisibilité et d'homogénéité. Aussi, nous nous félicitons de l'instauration d'une assurance vieillesse pour les aidants afin de reconnaître les efforts que ces personnes fournissent au quotidien et de leur ouvrir des droits sociaux spécifiques. L'AVA bénéficiera aux actuels bénéficiaires de l'assurance vieillesse des parents au foyer qui assument la charge d'un enfant ou d'un proche handicapé et sera par ailleurs élargie à d'autres publics, qui ne bénéficient pas aujourd'hui de la prise en compte de leur situation d'aidant, dans la constitution de leurs droits à la retraite : il s'agit des personnes qui ne cohabitent pas avec la personne dont ils assument la charge et avec laquelle ils ne présentent pas de liens familiaux étroits, ainsi que des parents d'enfants éligibles à un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

les associations représentant le secteur du handicap et de la perte d'autonomie sont très critiques par rapport à ce projet de loi. en discuter, mais vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous pensiez sûrement être entre vous, la droite réunie ... Mais non, nous sommes là, nous ne lâchons rien et nous ne lâcherons pas les Françaises et les Français mobilisés dans la rue contre ce projet.

À ce titre, le Collectif Handicaps a rappelé le caractère restrictif de l'extension aux seuls aidants des enfants handicapés percevant le complément à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, c'est-à-dire aux enfants dont le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 80 %. Notre amendement vise à réparer cette restriction. Il tend à proposer l'affiliation à l'assurance vieillesse des aidants aux parents dont l'enfant perçoit d'éducation de l'enfant handicapé inférieure à 50 %. Il n'est pas rare, en effet, que des enfants dans cette situation, même scolarisés à l'école ordinaire, ne puissent pas être accueillis toute la journée et tous les jours

L'élargissement de la possibilité de valider des trimestres à un plus grand nombre d'aidants prévue par l'article 12 est positive, certes, mais ces dispositions restent malheureusement trop restrictives et très en deçà de ce qui est attendu, au vu de la brutalité de votre réforme. Vous auriez pu faire davantage ! Cet amendement vise donc à élargir les critères d'affiliation à l'assurance vieillesse des aidants en l'ouvrant à tous les parents d'enfants handicapés ayant perçu une allocation d'éducation de l'enfant handicapé handicapé de base, et donc pas seulement à ceux qui sont éligibles à un complément, dans une logique d'ailleurs de simplification des démarches et de l'accès au droit. Comme c'est le Collectif Handicaps qui nous en avait parlé,

âgé ou handicapé, selon une étude publiée jeudi 2 février par la Drees. Particulièrement exposés au risque d'isolement et d'épuisement, ces 9,3 millions d'aidants familiaux mettent souvent leur vie professionnelle entre parenthèses. Pour qu'ils ne soient pas lésés au moment de la retraite, l'exécutif souhaite renforcer leurs droits avec la création d'une assurance vieillesse pour les aidants. À l'heure actuelle, 60 000 aidants bénéficient du dispositif de l'assurance vieillesse du parent au foyer. Selon l'étude d'impact, cette assurance vieillesse des aidants doit profiter à 40 000 nouveaux bénéficiaires. Le collectif interassociatif des aidants familiaux est satisfait de la reconnaissance de l'impact du rôle d'aidant sur les carrières, mais déplore un projet insuffisant : il s'agit d'une réécriture du dispositif existant, les droits sont identiques, ils sont les nouveaux. La vision des aidants est très orientée vers le handicap et ne prend pas en compte la situation des personnes malades ou âgées. Les associations d'aidants regrettent également la limitation de l'affiliation à l'assurance vieillesse des aidants. Notre amendement vise donc à étendre l'affiliation à l'AVA à tous les parents d'un enfant dont le taux d'incapacité est de 50 % et des parents d'un enfant en situation de handicap, dès lors qu'il est éligible à l'AEEH de base. Quel

le complément et l'affiliation à l'assurance vieillesse pour les aidants, c'est parce que l'attribution du complément est prévue spécifiquement quand l'aidant est tenu d'arrêter son activité professionnelle ou de la réduire à un point qui l'empêche de cotiser à l'assurance vieillesse classique.

toutes les procédures qu'offrent la Constitution et le règlement, en espérant certainement que nous nous lasserions et que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. La droite sénatoriale sur cette question des retraites

Cet amendement vise à ce que les décisions réglementaires en matière d'incapacité d'enfant ou d'adulte nécessitant la présence d'un aidant soient accompagnées d'un éclairage des instances représentatives des personnes en situation de handicap. Selon le baromètre 2017 de la fondation April, en partenariat avec BVA, 11 millions d'aidants familiaux, soit un Français sur six, accompagnent au quotidien un proche en situation de dépendance en raison de son âge, d'une maladie ou d'un handicap. Ces chiffres sont en constante augmentation. En 2030, selon les projections, un actif sur quatre sera aidant. Selon ce même baromètre, 54 % de ces personnes aidantes ignorent encore leur statut d'aidant. L'affiliation à l'assurance vieillesse permet à l'aidant familial de valider des trimestres pour sa retraite, sans qu'il ait besoin de verser des cotisations auprès de cette caisse. Par ailleurs, des diagnostics largement convergents montrent qu'il est nécessaire de mettre en place un véritable statut du proche aidant, un statut qui lui confère un certain nombre de droits plus complets et mieux identifiés, notamment en matière de cotisations à la retraite. Il s'agirait de revoir quel taux d'incapacité permanente d'un enfant ou d'un adulte nécessite son accompagnement au quotidien par ces aidants. Cette proposition est de bon sens. Nous demandons simplement la consultation des instances

Breuiller. Cet amendement vise à garantir que l'intention du législateur sera respectée sur ce sujet important. Après avoir refusé d'écouter les organisations syndicales, après avoir utilisé le 47-1, le Gouvernement recourt, de façon excessive selon nous, à des décrets. Compte tenu de l'importance du décret mentionné ici et des difficultés de prise en compte du point de vue des acteurs concernés, il nous semble indispensable, à mes collègues de groupe et à moi-même, que le Conseil d'État soit associé à la rédaction de ce décret.

le droit d'amender et leur laisse celui de soliloquer ? « Auriez-vous décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement ? « Espériez-vous que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées ? Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas. »

Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus : nous ne lâcherons rien, nous ne les lâcherons pas. Ma deuxième demande de rapport porte sur la lisibilité du système et sur le taux de non-recours au dispositif prévu à l'article 12 de ce projet de loi.

Celui-ci s'explique de différentes manières : non-connaissance de l'accès à ces prestations, complexité administrative, méfiance envers les administrations ou encore abandon de la demande à cause de la longueur des procédures. En France, depuis la dématérialisation des prestations sociales, l'accès aux droits s'est complexifié, en particulier pour les personnes en situation de précarité. Le non-recours à l'assurance chômage, par exemple, a atteint 30 % en 2018-2019, ce qui signifie qu'environ 540 000 personnes éligibles à l'assurance chômage n'en bénéficiaient pas. pas. C'est un problème qu'il faut prendre en charge. Alors que l'article 12 du projet de réforme du Gouvernement prétend faciliter la lisibilité de l'accès aux droits, notamment pour les aidants, la création d'une assurance vieillesse des aidants, nous sommes en droit de nous demander si ce nouveau dispositif ne va pas encore entretenir le flou sur les modalités d'accès à ces prestations. Il est plus qu'urgent de mettre en place des solutions concrètes contre le non-recours, comme l'automatisation des prestations sociales, qui permettrait aux Français de recevoir les prestations auxquelles ils ont droit sans en faire la demande. C'est pourquoi notre groupe parlementaire demande un rapport sur les conséquences de ce nouveau dispositif sur la lisibilité du système d'assurance vieillesse. Je vous rassure, monsieur le ministre, vous n'aurez pas besoin de vous lever pour me donner un avis favorable sur cette proposition, puisqu'il s'agit d'une demande de

le sort qui est réservé ici à ce genre d'amendement, d'autant que vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites réunies et coalisées ici, mais nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas. L'AVA, cette assurance vieillesse des aidants, exclura donc les parents des enfants handicapés dont le taux d'invalidité est inférieur

à l'aide des proches des enfants handicapés. La place croissante des aidants dans nos débats n'est peut-être que le revers de la médaille d'une politique inclusive qui ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Il est facile d'invoquer l'inclusion à l'école, au travail ; il semble beaucoup plus difficile à l'État de doter l'éducation nationale d'auxiliaires d'éducation formés et en nombre. formés et en nombre. Le recours aux aidants familiaux dans un contexte d'inégalité salariale entre les femmes et les hommes n'est alors que la persistance d'un modèle patriarcal où la charge du soin est supportée

pour nous faire l'écho de leur colère contre cette réforme, que le Gouvernement veut nous imposer à marche forcée en bâillonnant le Parlement et en usant pour cela de toutes les procédures que lui accordent le règlement et la Constitution. Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas.

dans un cadre non professionnel, à une personne handicapée ou à une personne âgée dépendante. J'en profite pour saluer le travail précieux réalisé par mon camarade Pierre Dharréville, député des Bouches-du-Rhône, pour sa proposition de loi

comprendriez : « Vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien. Nous ne les lâcherons pas. » Je confirme le message de Mélanie Vogel et je vous envoie le même. Notre système de retraite ne tient pas suffisamment compte du travail du,

ses parents, qui passe l'aspirateur pour que d'autres n'aient pas à le faire. Ce travail n'offre pas de droits à la retraite. Au contraire, la personne qui va passer une partie de sa journée à faire ce travail a forcément moins de temps et moins d'énergie disponible pour des activités salariales.

aide entraîne une diminution de leur revenu annuel moyen. En effet, le revenu reconnu pendant ces périodes étant considérablement inférieur, il tire le revenu annuel moyen vers le bas et l'aidant se retrouve avec moins de droits à la retraite. Cet amendement vise donc à demander au Gouvernement un rapport pour évaluer la possibilité d'exclure ces années du calcul du salaire annuel moyen, et ce même si vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement.

En effet, seul un membre de la famille peut bénéficier de la majorité des trimestres et l'aidant doit cesser totalement de travailler pendant une période de trente mois, éventuellement interrompus, pour toucher les trimestres majorés. Par ailleurs, certains aidants n'entrent dans aucune case et ne bénéficient d'aucune aide. Ainsi, un aidant dont le parent est malade du cancer ne bénéficie ni d'un congé de proche aidant ni de droits à la retraite. Avec votre réforme, le nombre d'aidants affiliés à l'AVA

pour les aidants à deux ans au lieu d'un an actuellement. Je vais terminer par une petite répétition dans les règles de l'art. Dans la mythologie grecque, Sisyphe est condamné à faire rouler un rocher en haut d'une montagne jusqu'à la fin des temps, puisque ce rocher finit toujours

par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien la commission ?

dont les besoins de main-d'oeuvre fluctuent énormément sur une année complète. La situation de ces travailleurs, qui connaissent une précarité inhérente à des professions rythmées par les saisons, est loin d'être satisfaisante, en matière tant de salaire que de conditions de travail.

Le COR a rappelé, dans son dernier rapport annuel, que, si des progrès ont été réalisés ces dernières années en matière d'emploi des seniors, la question des transitions vers la retraite reste prégnante, car une proportion sensible des assurés passent par des périodes de chômage ou d'inactivité entre leur sortie définitive du marché du travail et leur départ à la retraite. Par rapport au nombre de personnes en situation de cumul emploi-retraite, le dispositif de retraite progressive reste, selon les termes de la Drees, très marginal. Pourtant, les bénéfices de la retraite progressive pour la santé sont nombreux, puisque des chercheurs ont noté, entre autres bienfaits, une réduction de la fatigue et du stress, sources de risques psychosociaux. Il nous semblerait juste et attractif pour le dispositif que les bénéficiaires de la retraite progressive puissent jouir de leurs droits à la retraite sur la base d'un temps plein. temps plein. Vous pourriez aussi décider de retirer cette réforme qui va, nous le savons, prolonger le sas de précarité de milliers de personnes supplémentaires, sans emploi ni retraite. La Drees révélait en 2020 que le taux de pauvreté des personnes « ni en emploi ni en retraite » de 53 ans à 69 ans était de 32 %. Est-ce cela, monsieur le ministre, que vous signifiez par « Faciliter les transitions entre emploi et retraite » ? Faciliter pour qui ? Pas pour les classes populaires ni pour les plus vulnérables. Et je ne voudrais pas que l'on oublie que vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions les retraites des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes

à la fonction publique et aux indépendants. Nous trouvons regrettable de ne pouvoir échanger sur ces deux outils nouveaux, puisque vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas Je reviens à l'article 13. La libéralisation du dispositif cumul emploi-retraite vise à faire travailler les retraités ayant une pension de retraite insuffisante. Le but affiché est de mettre un peu de beurre dans les épinards de ceux et celles qui ont travaillé dur et qui n'en peuvent déjà plus. Le cumul emploi-retraite est inégalitaire. Seules sont concernées les personnes qui disposent de qualifications reconnues durant leur carrière, qui partent en bonne santé, avec des pensions déjà correctes, et qui peuvent reprendre facilement une activité. Au lieu de corriger les inégalités de carrière, notamment l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, cet article risque de fragiliser encore davantage la santé des personnes qui vont devoir poursuivre une activité salariée au-delà de 64 ans. Avec vos deux années de travail obligatoire, les personnes qui auront des carrières pénibles ne pourront plus travailler comme vous le leur demandez. Par exemple, dans les Côtes-d'Armor, mon département, que peuvent bien penser les ouvriers, les ouvrières, les aides à domicile sur le dispositif de cumul emploi-retraite, alors qu'ils sont déjà cassés à 45 ans ? Je puis vous dire qu'ils n'aspirent pas à ce cumul. Ils attendaient

des mesures aux philosophies opposées. D'un côté, il favorise et améliore le recours à la retraite progressive, qui permet aux travailleurs de partir à 60 ans, offrant aux seniors une transition vers la retraite en réduisant leur temps de travail, sans

des employeurs de souvent préférer les ruptures conventionnelles à ce dispositif de maintien dans l'emploi des seniors. Ainsi, en 2020, seuls 23 800 salariés bénéficiaient d'une retraite progressive. D'un autre côté, cet article 13 ouvre des droits pour les retraités qui décideraient de reprendre le travail en ayant recours au cumul emploi-retraite. Cette disposition aurait dû être précédée d'un débat sur la société que nous voulons. Voulons-nous une société où nos anciens

travailler. Il faut bien avoir en tête qu'il s'agit non pas de retraités qui souhaitent reprendre une activité professionnelle, mais bel et bien de retraités qui n'ont pas d'autre choix financièrement. La parole Breuiller, sur l'article. La retraite progressive est un dispositif qui pourrait être efficace pour faciliter la transition vers la retraite, surtout pour les emplois les plus difficiles, même si nous jugeons que le Gouvernement ne va pas assez loin pour démocratiser et améliorer ce dispositif qui est loin d'être parfait. En effet, les retraités ne s'en saisissent pas assez puisque seulement 2 % d'entre eux le font. Cet article vise à changer la donne en ouvrant ce dispositif aux fonctionnaires et en imposant aux employeurs de justifier leur refus quand un salarié en fait la demande. Nous proposons, pour notre part, de rendre impossible pour l'employeur le refus d'une telle demande : cela devrait donc devenir un véritable droit. Le problème avec ce dispositif, c'est qu'il aurait fallu maintenir cette possibilité de départ à la retraite progressive à 60 ans, voire plus tôt pour les carrières longues.

pas le montant de leur retraite. Bien que la retraite progressive soit un élément très utile pour faciliter la transition vers la retraite, nous ne pouvons nous résoudre à voter ce dispositif ... Heureusement, nous n'aurons pas à le voter, puisque vous avez choisi

Ce ne sera pas le cas. Et même si on ne peut plus débattre, même si nos amendements ne sont pas votés, nous pouvons toujours- je vous en remercie, monsieur le président, de l'avoir souligné -les retirer. Je signale au Gouvernement qu'il a aussi le droit de retirer son projet de réforme

Ces petits points de PIB reposent sur les travailleurs et sur l'augmentation sans fin de leur temps de travail. Dans la poursuite de cette logique sans fin, nous discutons donc d'un article qui vise à favoriser le cumul emploi-retraite pour, même à la retraite,

de précarité. J'aurais aimé développer mon propos, mais j'ai reçu à l'instant un message de Joël Labbé, qui me demande de vous lire le message

des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien, et nous ne les lâcherons pas ! Quel est l'avis de la

qui consiste à faire travailler tout le monde plus longtemps, y compris à partir du moment où les personnes liquident leurs droits à la retraite. Notre conception de la société est à l'opposé : nous souhaitons que la retraite permette de profiter de la vie sociale, familiale, culturelle et sportive, de s'émanciper, de bénéficier du droit au repos et au temps libre.

illégitime. Et quelle que soit l'issue de son examen, la bataille pour son retrait se poursuivra. Je vous le dis, nous ne lâcherons pas, nous continuerons à soutenir le peuple qui est dans la rue et qui manifeste pour ce retrait, et nous sommes nombreux !

rapporteur. Cet amendement vise à préciser que l'estimation indicative globale (EIG), adressée tous les cinq ans aux assurés à partir de 55 ans, inclut également des informations sur les règles applicables aux fonctionnaires en matière de cumul emploi-retraite.

Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons pas ! Le présent amendement vise à mettre au jour l'inégalité du dispositif de cumul emploi-retraite. Pour de nombreuses personnes qui craignent de ne pas pouvoir

De plus, le cumul emploi-retraite est un dispositif profondément inégalitaire, car il s'adresse essentiellement aux personnes qui disposent de qualifications reconnues durant leur carrière, qui partent à la retraite en bonne santé, qui touchent une pension correcte

Alors que l'article 13 vise à rendre le cumul emploi-retraite créateur de droits, nous pensons que la priorité est plutôt de corriger les inégalités de carrière, qui concernent particulièrement les femmes, et d'augmenter le montant des pensions.

ne contient en aucun cas des mesures qui amélioreront le quotidien des Français, bien au contraire. Il faut conclure ! Son but est de pousser les Français les plus précaires à travailler plus longtemps l'intégration du dispositif de cumul emploi-retraite. La parole est

que vous offrent la Constitution et le règlement. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien et nous ne les lâcherons pas !

comme vous le demandez. Nous aurions souhaité une loi Travail portant sur l'emploi des seniors et le vieillissement au travail. L'adaptation des conditions de travail à la fin de la carrière aurait dû être votre priorité Nous ne le répéterons jamais assez : agir sur le taux d'emploi des seniors et l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sont des solutions pour le financement

essentiellement aux personnes qui disposent de qualifications reconnues durant leur carrière, qui partent en bonne santé avec des pensions correctes et qui, à ce titre, peuvent reprendre plus facilement une activité. Selon l'Insee, les bénéficiaires actuels du cumul emploi-retraite sont ainsi majoritairement des personnes qui qui ont une carrière complète ou un niveau de pension supérieur à la moyenne. Plutôt que de corriger les inégalités de carrière, qui concernent particulièrement les femmes, cet article risque de fragiliser encore davantage les personnes qui devront poursuivre une activité salariée au-delà de 64 ans. Celles et ceux qui ont recours au cumul emploi-retraite sont également celles et ceux qui travaillent au-delà de 62 ans pour bénéficier de la surcote. Ce sont les salariés dont la rémunération ne permet pas de percevoir une retraite digne et qui doivent trouver des solutions pour avoir une pension suffisante et faire face à la hausse des prix du quotidien ainsi qu'au coût des soins non remboursés par la sécurité sociale. Voilà encore un amendement qui ne pourra pas avoir de suite puisque vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution et le règlement du Sénat. Vous espériez sans doute que nous laisserions la retraite des Français entre les mains des droites coalisées. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. Nous ne lâcherons rien, et nous ne les lâcherons

collègues, vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent Vous espériez sans doute que nous laisserions les retraites entre vos mains. Nous ne sommes pas dupes, les Français non plus. En effet, nous ne lâcherons rien, absolument rien

rien ! Le Gouvernement propose de modifier le dispositif de cumul emploi-retraite en permettant l'acquisition de nouveaux droits à pension, lorsque ce cumul est réalisé après le départ à taux plein et après liquidation de toutes les pensions. Cette mesure peut apparaître comme une bonne chose, monsieur le rapporteur, en ouvrant des droits pour celles et ceux qui reprennent une activité professionnelle. Or, aujourd'hui, le cumul emploi-retraite s'adresse essentiellement à celles et à ceux qui ont exercé les métiers les moins pénibles. Surtout, en prévoyant l'ouverture de droits dès lors que les salariés disposent d'une carrière complète, on oublie tout de même un peu les femmes En effet, les emplois à temps partiel sont occupés à 80 % par des femmes, dont la carrière est hachée du fait d'interruptions. Elles sont environ 20 % à attendre l'annulation automatique de la décote à 67 ans

nous ne sommes absolument pas contre les dispositifs de transition, bien au contraire ! Ce que nous dénonçons, ce sont les systèmes subis : temps partiel subi et cumul emploi-retraite

Oui, mes chers collègues, vous avez décidé de dévitaliser la fonction parlementaire par l'addition de toutes les procédures que vous offrent la Constitution

Nous ne lâcherons pas non plus le débat sur l'hypocrisie des mesures que vous présentez comme des pseudo-avancées. C'est le pâté de cheval et

progressive pouvait rendre difficile l'accès à une carrière complète. Je tiens à bien préciser que lorsque l'on est dans un système de retraite progressive et que l'on continue à travailler à temps partiel tout en ayant liquidé partiellement sa pension de retraite, on continue à cotiser.